la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. J'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat : le respect- respect des uns et des autres, mais aussi celui

et indépendants. Monsieur le Premier ministre, un maire bâtisseur, c'est, pour nos concitoyens, un maire bétonneur. Voilà la sentence qu'entendent aujourd'hui nombre de maires qui ont choisi, notamment en zone tendue, de se saisir à bras-le-corps de l'épineuse question du logement.

Alors que s'est ouvert, hier, le Congrès des maires- occasion pour moi de saluer les nombreux élus présents dans notre beau Sénat -, la question du logement apparaît comme centrale sur notre territoire national. Il est plus que jamais nécessaire de porter un discours politique offensif, seule façon de réhabiliter l'acte de construire dans les zones où l'offre de logement est inférieure à la demande. Cette question est au coeur des préconisations de la commission pour la relance durable de la construction de logements, présidée par François Rebsamen et qui a remis récemment le tome II de ses conclusions. La commission, dans ses premières conclusions, recommandait aux élus d'affirmer qu'une densité heureuse était possible, à condition de veiller à la qualité des logements et des espaces urbains. Ce discours politique doit bien évidemment s'accompagner de mesures financières concrètes de soutien aux communes et intercommunalités. Des mesures ont déjà été prises dans le cadre du plan de relance. Ainsi, 1 288 communes ont reçu 142 millions d'euros, pour plus de 67 000 logements construits

de contractualisation recentré sur les territoires tendus où l'offre de logement fait défaut, tout en optimisant le foncier disponible au regard de sa rareté et de son coût. Les intercommunalités et communes des zones tendues sont les premières intéressées et doivent s'engager fortement sur des objectifs de production de logements neufs. Monsieur le Premier ministre, au moment où les élus de notre pays ont rendez-vous à Paris, pouvez-vous confirmer à la représentation nationale les termes de cette contractualisation ainsi que ses modalités sur un sujet, le logement, qui doit mobiliser toutes les énergies ? La

de partager avec vous toutes et vous tous le diagnostic suivant : la situation du logement dans notre pays est préoccupante. Nous pourrions passer du temps à identifier les causes de cette situation.

la décision de moins construire de logements- notamment dans de grandes agglomérations. Je le dis : cela est sans doute regrettable. Néanmoins, il ne s'agit pas de la seule raison à cette situation ; nous pouvons en convenir. J'ai souhaité, en lien avec la ministre déléguée chargée du logement, Mme Emmanuelle Wargon, prendre un certain nombre de dispositions pour essayer de faire face à cette situation, qui intéresse la vie quotidienne de nos concitoyens. Vous l'avez rappelé, j'ai d'abord demandé à une commission

Je me permets de vous les rappeler rapidement, puisque vous en avez cité quelques-unes. Il s'agit tout d'abord de la contractualisation dans les zones tendues. Vous le savez, dans ce domaine comme dans d'autres, je crois au contrat, avec le représentant local de l'État, le préfet, et le président de la métropole, de l'agglomération ou de la ville

Il est prévu dans le projet de loi de finances la compensation intégrale par l'État de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant dix ans pour les logements sociaux agréés en 2021 et jusqu'à la fin de l'actuel mandat..

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, « déserts médicaux » : cette expression est devenue le symbole d'un sentiment profond de relégation- en secteur rural, mais aussi en ville. La question s'était imposée dans le grand débat alors que cette urgence n'avait pas été jugée prioritaire par le Président de la République. Renforcée par la crise sanitaire, l'inégalité d'accès aux soins fait aujourd'hui partie des premières préoccupations de nos concitoyens. Cette inégalité n'est pas du seul fait de votre gouvernement, monsieur Castex. C'est certain. Mais il faut que chacun se mobilise pour la résorber. Je salue les nombreux élus locaux présents dans ces tribunes à l'occasion du Congrès des maires. Ils sont, chaque jour, sur le terrain et luttent contre une telle désertification.

Ce dispositif, adopté contre votre avis, monsieur le Premier ministre, mais promulgué par le Président de la République le 24 juillet 2019, attend toujours son décret d'application. La procrastination du Gouvernement sur ce sujet est coupable : coupable, car vous n'appliquez pas la loi qui a été votée ; coupable, car vous abandonnez, de fait, des millions de Français et leurs représentants à leur sort. En mai dernier, M. Taquet n'avait rien répondu à la même question posée ici même par Bernard Jomier. Vendredi dernier, sur l'interpellation du président Retailleau dans cet hémicycle, M. Taquet renvoyait l'éventuelle publication de ce décret au mois de mars. Toutefois, rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, nous vous demandons une réponse claire, un calendrier précis.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président Kanner, j'ai déjà eu l'occasion à de multiples reprises de m'exprimer, y compris devant le Sénat, sur le problème de la désertification médicale,

extrêmement malthusien depuis des décennies ! Cela vous dérange peut-être, mais c'est la vérité absolue : absolue ! Voyez-vous, monsieur Kanner, vous étiez aux affaires jusqu'en 2017

qu'il manque de médecins dans ce pays ! Et l'on voudrait nous faire croire que la publication d'un décret va y remédier ! Bien sûr que non, monsieur le sénateur, bien sûr que non ! À qui ferez-vous croire cela ? Je sais bien que nous sommes en période électorale, mais vous ne nous ferez pas prendre des vessies pour des lanternes

Madame la ministre, je profite de cette semaine spéciale pour le Sénat- marquée par l'accueil de nombreux élus locaux à l'occasion du Congrès des maires et présidents d'intercommunalité -pour vous interroger sur le sujet hautement sensible de la cybersécurité, qui touche le secteur privé, mais aussi les collectivités territoriales. L'attaque de plusieurs grandes villes a fait la une des journaux ces derniers mois : je pense notamment à La Rochelle, Évreux ou encore Bayonne. Mal informées et mal armées, elles ont pour certaines été perturbées, voire paralysées pendant des semaines. les petites communes sont encore plus vulnérables, par manque d'ingénierie et de services dédiés. Dans mon département, la commune de Surat, dotée de moins de 600 habitants, a été victime d'un rançongiciel, qui a bloqué l'accès à toutes les données et réclamé le paiement d'une rançon pour le rétablir. D'après D'après une étude, en 2020, au moins 4 % des communes françaises ont été piratées et 14 % des victimes de rançongiciels étaient des administrations. Du fait du recours massif au télétravail et à la dématérialisation, la crise sanitaire a démultiplié les cyberattaques et rendu encore plus vulnérables nos collectivités locales. Dans le cas de Surat, la communauté d'agglomération, disposant de l'ingénierie nécessaire, a proposé un groupement de commandes pour le seul audit des installations informatiques, qui a coûté plus de 30 000 euros, sans aucun financement. Or le Gouvernement a annoncé en février la mobilisation de 1 milliard d'euros pour une stratégie nationale de cybersécurité, dont une partie doit être consacrée aux administrations. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur l'utilisation de cette enveloppe ? Les données en jeu sont particulièrement sensibles : sécurité sociale, état civil, informations bancaires ou médicales. Les conséquences peuvent être lourdes, y compris sur le plan de l'image. Nous savons que cette méthode est de plus en plus utilisée à des fins de déstabilisation politique. Les collectivités ont besoin d'accompagnement, car elles n'ont souvent pas les compétences humaines et techniques nécessaires, dans un domaine qui évolue constamment. Aussi, madame la ministre, que peut-on faire pour mieux informer et mieux accompagner les élus face à ces nouveaux dangers ? La parole est à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le sénateur Éric

qui font la force de notre République. Vous l'avez dit, nous faisons face à une augmentation très forte des cyberattaques visant nos collectivités territoriales.

et des communications électroniques, Cédric O, l'État accompagne les collectivités territoriales pour renforcer leur sécurité informatique. Dans chaque région, un référent de l'Anssi est chargé de conseiller les collectivités et de répondre à leurs questions. cybermalveillance.gouv.fr recense l'offre locale de services de sécurité informatique que peuvent mobiliser les collectivités territoriales. Dans le cadre de France Relance, un parcours de cybersécurité est proposé aux collectivités territoriales, comprenant notamment un accompagnement opérationnel effectué par des prestataires spécialisés. Nous avons invité toutes les associations d'élus à informer leurs membres de l'existence de ce dispositif, dont plus de 500 collectivités ont déjà profité. De manière plus générale, l'État a mobilisé plus de 700 millions d'euros de crédits du programme d'investissements d'avenir et de France Relance sur la thématique de la cybersécurité, dont une partie est dédiée

se tient en ce moment même le 103 Congrès des maires : celles et ceux, vous le savez, qui ont pour mission de gérer au quotidien les besoins de tous les Français. Ils le font au plus près du terrain, alors que l'État et les autres strates administratives, bien trop nombreuses, toujours en place malgré les promesses présidentielles, doivent assurer le fonctionnement libre, égal et fraternel de nos institutions et des projets structurant nos territoires et garantir la solidarité. « Nous réduirons le millefeuille administratif. Nous supprimerons au moins un quart des départements », avait dit Emmanuel Macron alors qu'il était en campagne. De ces promesses, que reste-t-il ? Depuis cinq ans, et particulièrement pendant la crise sanitaire encore en cours, vous avez vanté le couple préfet-maire, capable de miracles, de résoudre tous les problèmes, au plus près des citoyens, avec toute la puissance de l'État. Comment se satisfaire du pouvoir croissant du préfet dans la tenue des politiques publiques, et de cette prépondérance de la déconcentration aux dépens de la décentralisation ? Où sont coconstruction, coopération, concertation, quand en réalité les maires n'ont de cesse d'essayer de comprendre et d'adapter des décisions venues d'ailleurs, d'un pouvoir exécutif qui n'avait plus été aussi centralisateur depuis des décennies ? Interrogez les maires, vous serez édifiée. Interrogez les citoyens : vous savez, celles et ceux qui ne se déplacent plus

monsieur Benarroche, de travailler beaucoup avec Marseille. Je me tourne également vers d'autres sénateurs des Bouches-du-Rhône. À la suite de la visite du Président de la République à Marseille

Merci, madame la ministre. Néanmoins, au gré des lois, des amendements, des décrets et des ordonnances, vous refusez- souvent avec la droite parlementaire, d'ailleurs-de donner aux maires le pouvoir d'agir pour et avec leurs citoyens

La parole est à Mme Colette Mélot, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires.

Entre 700 000 et 1 million d'élèves en sont victimes chaque année. Derrière ces chiffres, une multitude d'enfants et d'adolescents font face à des insultes, des menaces, des coups, à un stress permanent, qui, parfois, mène au pire. Derrière ces chiffres, ce sont d'autres enfants qui se permettent, en dépit de toutes les règles du savoir-être, en dépit de la loi, de commettre des actes intolérables. La récente mission d'information sénatoriale, dont j'étais la rapporteure, propose des mesures concrètes pour endiguer la violence à l'école. L'une d'entre elles vise à faire du harcèlement scolaire une grande cause nationale pour 2022. La protection de la jeunesse à l'égard de toute violence mérite cette mobilisation générale. Quelle est, monsieur le ministre, la position du Gouvernement sur cette proposition ? Nous devons ériger des remparts plus efficaces contre la violence à l'école, développer une culture de la bienveillance, du courage et de la protection dans chaque établissement scolaire. contre le harcèlement à l'école, dont j'aimerais connaître, monsieur le ministre, le bilan. J'aimerais également savoir combien d'établissements sont engagés dans le dispositif depuis sa généralisation en septembre dernier. Frances Haugen alertait le Sénat la semaine dernière sur la brûlante nécessité de renforcer le. Nous devons mutualiser nos moyens pour obliger les plateformes à protéger leurs utilisateurs en investissant dans la sécurité et la modération des contenus, afin de rendre compatibles technologie et démocratie. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, est-il envisagé d'inscrire ce sujet parmi les priorités portées par la France ?

contre 10 000 ambassadeurs l'an dernier. Nous sommes donc concrètement en train de former des élèves à lutter contre le harcèlement, au quotidien, avec ces ambassadeurs. En outre, 237 formateurs académiques ont déjà formé 10 330 adultes. Ce chiffre évoluera de jour en jour, en vertu de la généralisation du programme dont je vous parlais. Cet après-midi, je rencontre les responsables des plateformes pour aller plus loin dans la lutte contre le cyberharcèlement- dans le sens que vous préconisez dans votre rapport. Je le répète, je suis en accord complet avec vos préconisations, et nous avancerons encore d'un cran dans ce sens. Il faut une unité nationale pour lutter contre ce fléau. La parole Je vous remercie, monsieur le ministre. La peur doit changer de camp pour que la jeunesse reste ce champ des possibles dans lequel chacun peut grandir et s'épanouir, dans le respect des valeurs qui fondent notre République.

qui a dit, à juste titre, que la situation du secteur de la construction neuve était préoccupante. Elle est plus que préoccupante, monsieur le Premier ministre, puisque- et ce n'est pas M. Denormandie qui me

à 20 000 ménages salariés, dans le cadre de l'avenant « relance » signé avec les partenaires sociaux. Nous travaillons en parallèle sur l'accès locatif ; nous ne restons pas les bras croisés sur ce sujet. Les propriétaires seront ainsi incités à proposer des loyers plafonnés dans le parc existant, grâce au dispositif « Louer abordable

Le concours Lépine des mesures attentatoires aux libertés publiques se poursuit donc inexorablement sur notre continent, étape après étape, sans que l'on se pose jamais la question d'une marche arrière.

Dans notre pays, plusieurs responsables politiques, et non des moindres, se sont positionnés en faveur de cette évolution. Vous-même, monsieur le ministre, qu'en pensez-vous ?

solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, je vous reconnais le mérite de la constance. Vous vous êtes prononcé systématiquement contre l'usage du passe sanitaire, parmi les outils disponibles pour lutter contre la diffusion du virus. Vous avez toujours été contre, vous l'avez dit, c'est votre conviction et vous êtes fondé à l'exprimer. Permettez au Gouvernement de faire également preuve de constance : celle qui consiste à prendre au bon moment les bonnes mesures pour freiner la diffusion du virus et protéger la population française.

Un homme est emprisonné depuis bientôt trois ans dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, à Londres. Son nom est Julian Assange. Ce journaliste australien de 50 ans est poursuivi par la justice américaine. Son crime : avoir publié 700 000 documents diplomatiques et militaires, qui ont dévoilé au monde entier les activités d'espionnage de Washington, mais aussi les crimes de guerre commis par les États-Unis sur des terrains d'opération tels que l'Irak, ou à Guantanamo. Nous apprenions également par ce biais, en 2015, la mise sur écoute téléphonique de trois présidents de la République française : Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ces faits sont évidemment d'une gravité extrême. Monsieur le ministre, ma question est double

le passé ; elles avaient alors jugé qu'il n'y avait pas lieu d'apporter une réponse favorable à son accueil en France, en raison d'éléments liés à la situation juridique et à la situation de fait de l'intéressé.

Notre pays, garant des valeurs universelles de liberté et de démocratie, s'honorerait d'accorder à Julian Assange l'asile politique, afin que celui-ci échappe à toute extradition vers les États-Unis et évite ainsi une peine de 175 années de prison.

Monsieur le Premier ministre, il y a quatre ans, ici même, le Président de la République promettait de faire de la politique des territoires une priorité pour ce quinquennat. Quatre ans après, le moins que l'on puisse dire est que la déception domine. Au Sénat, toutefois, nous faisons toujours preuve de pragmatisme et nous avons, sous l'égide du président Gérard Larcher, proposé

-du préfet de département la porte d'entrée de l'État territorial dans nos départements et renforcer le couple maire-préfet. Nous

finalité : agir au plus près de nos concitoyens. Sur l'ensemble des mesures fortes que nous avons proposées, notre philosophie est toujours la même : il s'agit de faire en sorte que les élus, singulièrement les maires, encore de la capacité de décider de l'avenir de nos communes et de répondre aux aspirations de nos concitoyens. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre : allez-vous répondre à l'audace sénatoriale concernant ce texte 3DS ou celui-ci n'est-il voué qu'à devenir un énième texte d'ajustement ? La parole

je ne peux préjuger des positions que retiendront les députés. J'ai cependant le sentiment qu'ils apporteront d'utiles enrichissements au texte dans un esprit de rigueur et de responsabilité identique à celui qui a présidé aux travaux du Sénat.

À l'appui de cette thèse, identifie deux dérives : l'antiracisme et la lutte contre l'homophobie. Il me semblait, jusqu'alors, que l'antiracisme et la lutte contre l'homophobie faisaient partie des valeurs universelles,

au titre des principes de la République- « Liberté, Égalité, Fraternité » -, et nous avons aussi beaucoup insisté sur la laïcité, car c'est le cadre qui permet l'épanouissement de ces principes.

Bien entendu, la lutte contre le racisme, le féminisme, la lutte contre l'homophobie s'intègrent complètement dans « Liberté, Égalité, Fraternité », je le dis très fortement. Je soutiens les professeurs qui opèrent cette transmission des valeurs, il n'y a aucun doute sur ce point.

Elle était d'abord victime de harcèlement raciste, lesbophobe, homophobe. Elle s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus d'entendre « sale métisse » et « sale lesbienne ».

Ce scénario coûterait, au minimum, plus de 20 milliards d'euros aux finances publiques, pourtant déjà bien mal en point. Il est vrai que le « quoi qu'il en coûte » permet toutes les audaces ! L'essentiel n'est pourtant pas là. Derrière cette proposition, on retrouve le dessein, porté depuis dix ans déjà, avec François Hollande puis avec Emmanuel Macron, d'étatiser notre système de santé. Comment peut-on croire encore que l'État, champion des déficits, pourrait se charger de nouvelles dépenses ? S'il était aussi bon gestionnaire, cela se saurait, et les Français n'auraient pas à supporter à la fois des impôts record et une dette qui ne cesse de se creuser.

! Faute de réformes et de moyens, l'État régule les dépenses de santé par la pénurie ; c'est cela la réalité à laquelle les patients sont aujourd'hui confrontés. Étatiser les dépenses de santé, c'est aller chercher comme remède la cause même de nos déboires. Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas qu'étatisation rime avec grande illusion, et monopole d'État avec déficit ? avec déficit ? La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, monsieur le sénateur, de me permettre de discuter d'un rapport que ni vous ni moi n'avons lu, mais qui est d'ores et déjà largement commenté. Ni vous ni moi ne l'avons lu, puisqu'il sort demain. Il fait

pour le groupe Union Centriste. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Alors que vient de s'achever la conférence internationale de Paris sur la Libye, Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de Mouammar Kadhafi, a présenté dimanche sa candidature à l'élection présidentielle libyenne. C'est un électrochoc pour le pays, qui ne parvient pas à se reconstruire. La chute du régime de Mouammar Kadhafi devait ouvrir une nouvelle ère, plus démocratique et plus prospère. Dix ans après, tous les espoirs ont été déçus. La Libye n'a cessé de vivre dans le chaos, livrée aux milices souvent instrumentalisées par des puissances étrangères. Néanmoins, depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu le 23 octobre 2020, à l'issue de la conférence de Berlin, un processus de sortie de crise semble se dessiner. Il a été confirmé, le 15 novembre 2020, par l'adoption de la feuille de route politique libyenne à Tunis et, le 10 mars dernier, par l'approbation du Gouvernement d'unité nationale de transition. La prochaine étape, décisive, est celle des élections présidentielle et législatives du 24 décembre prochain. La candidature du fils de Mouammar Kadhafi peut mettre à mal le processus politique libyen. Avec des conséquences directes pour la France. Ainsi, le refroidissement de nos relations avec l'Algérie nous force à survoler la Libye pour gagner le Mali ; si ce pays s'embrase de nouveau, cela ne sera plus possible. La stabilité de la Libye est aussi pour nous un enjeu migratoire et de sécurité, sans parler de la responsabilité de notre pays dans cet échec cuisant. Monsieur le ministre, selon vous, le processus politique libyen est-il en danger ? Si tel est le cas, quelle sera votre action pour le conforter ?

lors de la conférence internationale pour la Libye, qui a été initiée par le Président de la République et à laquelle participaient tous les acteurs, soit seize chefs d'État ainsi que des pays représentés par certains de mes homologues.

après dix années marquées par des migrations irrégulières, du trafic d'êtres humains, des flux irréguliers d'armes, des ingérences étrangères ; bref, des années de désastre.

plusieurs autres, ce qui montre que le processus est dans une phase positive, même si certains veulent le retarder et l'empêcher. Merci, monsieur le ministre, de votre réponse, mais la Libye est au coeur de nombreux enjeux stratégiques, notamment pour l'Europe. Durant la dernière décennie, le pays n'a pas su endiguer la violence et la guerre civile. Il est devenu, comme la Syrie, le théâtre d'une guerre par procuration et un enjeu de convoitises à la fois régionales et internationales. Monsieur le ministre, la France doit absolument rester vigilante quant à l'évolution du processus libyen.

Pourtant, le principe de l'autonomie financière des collectivités et celui de leurs ressources propres, qui constituent les bases de cette décentralisation, ne cessent d'être remis en question. Les déclarations d'amour du Président de la République et du Gouvernement envers les élus, renouvelées encore à l'occasion du 103 Congrès des maires, ne peuvent dissimuler un processus de concentration des ressources financières des collectivités entre les mains de l'État. Votre réforme de suppression de la taxe d'habitation ne laissera bientôt plus aux maires que les taxes foncières et un tiers de l'ancienne taxe professionnelle comme ressources à pouvoir de taux. Ce n'est pas une question accessoire, car c'est toute la démocratie locale qui sera, à terme, remise en cause. En outre, si l'on ne fait peser l'impôt local que sur les seuls propriétaires et entreprises, le lien fiscal entre les habitants et leurs territoires ne tient plus qu'à un fil. Vous nous direz que l'État sera là pour compenser intégralement chaque euro perdu, mais nous savons ce que vaut la parole d'un État qui est toujours revenu sur ses engagements. Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), censé assurer une équité entre territoires, est de plus en plus mal compris par les communes. Madame la ministre, allez-vous enfin enrayer ce processus délétère de recentralisation et de creusement des inégalités entre nos territoires ? La parole est à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la sénatrice,

de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Permettez-moi de vous dire très simplement que, comme le Président de la République s'y était engagé au début de son quinquennat, nous avons mis fin à la baisse des dotations. La dotation

des communes aux ressources modestes ne bénéficient pas de ce fonds autant qu'elles le devraient, parce qu'elles sont considérées comme globalement riches depuis leur rattachement aux intercommunalités. Madame la ministre, nous attendons une action forte et rapide de la part du La parole est à M. Lucien Stanzione, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. et Républicain. Madame la ministre, fermeture de classes, fermeture de bureaux de poste, de trésoreries ou d'établissements de santé comme celui de Roquefraîche dans le Vaucluse ... Le Gouvernement opère une véritable casse du service public Alors qu'il s'était engagé à ne fermer aucune classe et aucune école rurale sans l'accord du maire à la rentrée de septembre dernier, la trajectoire observée est bien différente. La collaboration avec les collectivités territoriales semble avoir été délaissée au profit d'une application froide du seuil d'élèves, qui ne prend pas en compte la réalité de nos territoires. Dans le Vaucluse, trente-trois fermetures de classes sont à déplorer dont trois à Apt, dans un territoire qui La réduction des horaires d'accueil, voire la fermeture des bureaux de poste, comme à Robion, sont les signes de l'absence totale de considération des usagers. La fermeture des trésoreries publiques, comme à Langon, Paimpol ou encore Vaison-la-Romaine, et la suppression de 5 700 lits d'hôpitaux en pleine pandémie sont d'autres exemples. Face à toutes ces disparitions, la seule réponse que vous apportez est la dématérialisation et la création de quelques maisons France Services, en sollicitant financièrement les collectivités locales. Cette conception d'une société tournée uniquement vers les hyperconnectés et la concentration des services, sans considération de nos aînés, par exemple, n'est pas la nôtre. Madame la ministre, expliquez-nous comment vous ferez pour répondre concrètement aux besoins quotidiens des usagers

je ne peux pas vous laisser dire cela. Depuis 2017, de manière constante, ce gouvernement- il le fera encore en 2021, et encore en 2022 -remet des agents publics sur le terrain, des policiers, des greffiers ou des enseignants. Il n'y a jamais eu autant d'enseignants dans le premier degré qu'en 2022 ! Nous rouvrons des postes d'agents dans les préfectures et les sous-préfectures, alors qu'entre 2010 et 2017, sous

Madame la ministre, le service public est l'amortisseur de la crise. Il est l'engagement de la Nation au profit de ses concitoyens. Il garantit aussi l'égalité sociale. Ce sont les publics les plus fragiles qui subissent la disparition des services de proximité.

Monsieur le ministre, au moment même où se déroule le Congrès des maires et que mes collègues élus ultramarins nous partagent les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs territoires respectifs sur l'application de l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers, et alors même que les Antilles et la Guyane sont confrontées à des grèves, barrages routiers, manifestations et défilés, qui perturbent grandement la vie et l'activité économique de leurs habitants, il m'est d'avis qu'une solution pérenne prenant en compte la spécificité de ces territoires, souvent petits et déjà soumis à des pénuries de personnel en temps normal, doit être trouvée afin de répondre de manière décente à la prise en charge sanitaire des populations. Donner l'assaut à des personnels soignants ou aux pompiers, comme nous avons pu le voir sur les réseaux sociaux, ne peut être une réponse ; tout comme le report en Martinique ne résout pas le problème. Depuis quatre jours, une note de service du centre hospitalier de Saint-Martin, qui a largement circulé sur l'île fait part d'une réorganisation interne proposée par la direction. L'activité opératoire est très limitée, le service de chirurgie est fermé et le bionettoyage est assuré par un prestataire extérieur, alors même que l'hôpital est déjà fortement endetté. endetté. Les Saint-Martinois craignent de se rendre à l'hôpital, tant ils sont conscients de la dégradation de la prise en charge. Dans la population, on n'ose plus appeler le 18, car on ne sait pas si l'on aura une réponse. Assignations et réquisitions des pompiers montrent leur limite. Monsieur le ministre, dans le cadre de la différenciation et de nos spécificités ultramarines, une adaptation de la loi sur l'obligation vaccinale faite aux sapeurs-pompiers et aux soignants me semble indispensable. En effet, si le rôle de l'État de protéger la population contre la covid-19, il doit également assurer une couverture sanitaire décente de nos territoires. Protéger de la covid-19, oui

y compris dans les domaines les plus stratégiques. Je pourrais citer les médicaments ou les composants électroniques, mais je vais prendre un exemple dont on parle beaucoup moins, celui de notre agriculture. Depuis le début de l'année, nous assistons en Europe et particulièrement en France, à un triplement du prix des fertilisants indispensables à la croissance des cultures végétales sur tous nos territoires. Cette situation fait peser un grand risque économique et social à notre pays, qui doit faire face à un surcoût estimé à plus de 4 milliards d'euros. À cela s'ajouterait une pénurie d'azote, qui représente un véritable danger pour notre souveraineté alimentaire. Les productions accuseraient une diminution de leur teneur en protéines, tandis que les rendements seraient fortement affectés. Cette inquiétante hausse des prix prend notamment sa source dans une flambée des prix du gaz naturel, indispensable à la fabrication de l'azote, et qui est presque intégralement importé. Elle est amplifiée par l'existence de barrières tarifaires européennes sur les importations de fertilisants, dont des droits de douane et des taxes antidumping. Dans ce contexte, monsieur le Premier ministre- et vous aussi, monsieur le ministre de l'agriculture et de Nous avons perdu des pans entiers de notre industrie ; en sera-t-il de même pour notre agriculture ? Aussi, à l'aube de la présidence française de l'Union européenne, pouvez-vous décrire, ici, devant la représentation nationale, ce que vous comptez faire au niveau des instances européennes pour éviter ce cataclysme annoncé

La séance est suspendue. La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école est parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, avec ce second projet de loi de finances rectificative pour 2021, le Gouvernement tient d'abord ses engagements en faveur du soutien à l'économie et aux publics les plus touchés par la crise.

Je pense aux prêts garantis par l'État, prolongés jusqu'au 30 juin 2022, comme l'a annoncé le Président de la République. Près de 700 000 entreprises en ont bénéficié, pour un montant total engagé- donc garanti -de 141 milliards d'euros.

leur activité. L'équivalent de 3,6 milliards d'euros d'échéances fiscales a été reporté, permettant aux entreprises de reprendre leur souffle et de préserver leur trésorerie. Par ce soutien massif aux entreprises, le Gouvernement a voulu maintenir l'activité et l'emploi, et préserver les compétences, dans un effort inédit de lutte contre le chômage de long terme.

Au regard du chemin que nous avons parcouru, nous pouvons être collectivement fiers des résultats de notre action menée de concert : l'économie a été protégée avec succès et nous savons que, dans ces circonstances, Dorénavant, la situation a évolué et nous sortons pas à pas de la crise, même si nous savons bien que l'épidémie n'est pas éteinte et que l'incertitude continue de planer en matière sanitaire. En revanche, nous savons qu'en matière économique et sociale nous sortons de cette période de crise. En conscience, nous avons fait le choix de la précaution et du réalisme pour sortir progressivement des dispositifs d'urgence. Ainsi, dès l'été 2021, les dispositifs du fonds de solidarité, d'exonération de cotisations sociales et d'activité partielle ont été recentrés vers les entreprises les plus en difficulté.

Dans le projet de loi de finances rectificative que je vous présente, nous poursuivons cet effort. Ainsi, nous nous sommes engagés pour préserver le pouvoir d'achat des Français face à l'inflation, grâce à la mise en place de l'indemnité inflation annoncée par le Premier Par cette mesure exceptionnelle, nous visons un objectif de simplicité et de rapidité de mise en oeuvre, pour répondre le plus efficacement possible à la hausse des prix. C'est une mesure simple et rapide, en un mot, efficace, qui permettra à tous nos concitoyens- salariés, indépendants, retraités, chômeurs, allocataires des minima sociaux ou encore étudiants boursiers

de la crise. En prenant du recul sur les épisodes que nous avons traversés, je souligne d'abord que la stratégie économique du Gouvernement a rendu possible le rebond économique massif de notre économie et, par conséquent, la réduction du poids du déficit et de la dette par rapport à notre PIB.

Nos engagements en faveur du redressement des finances publiques se poursuivent encore au-delà, puisque, comme je l'ai indiqué, nous vous proposons d'annuler plus de 2 milliards d'euros de crédits de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », conformément à notre calendrier de sortie progressive des aides

L'exécution des dépenses sera conforme au niveau prévu dans la loi de finances initiale, à l'exception de quelques compensations de pertes de recettes liées à la crise sanitaire. Il s'agit par exemple de la dotation de 2 milliards d'euros que nous vous proposons d'accorder à France compétences.

En définitive, je crois que notre action a porté ses fruits. Grâce à l'effet conjoint de la révision à la hausse de la croissance, de l'annulation des surplus des crédits d'urgence et de la maîtrise des dépenses ordinaires,

Nous respecterons aussi notre objectif d'un déficit limité à 5 % en 2022, tel que nous l'avons annoncé lors de l'examen du programme de stabilité. De même, nous estimions au printemps dernier que notre dette atteindrait 117,8 % du PIB en 2021

continue à garantir la protection des Français, à favoriser la relance de l'économie et à préparer l'avenir pour que la France reste à la pointe dans ses domaines d'excellence. Ce texte prévoit la sortie progressive des dispositifs de soutien financier déployés pendant la crise. davantage sur les acteurs qui en ont le plus besoin et privilégie les politiques qui nous paraissent les plus efficaces. Il se prémunit du danger important que ferait courir la cessation brutale des mesures de soutien face à la crise. Nous devons veiller à toujours maintenir et accompagner la croissance, qui sera, je le répète, la clé du redressement des comptes publics, mais aussi celle de la relance et de la sortie de crise. Je pense que ces choix sont logiques et cohérents.

devrait en principe se contenter, comme à chaque fin d'exercice, de tirer les conséquences de l'année écoulée et de proposer un schéma de fin de gestion. Pourtant, dès son dépôt, ce texte ne se réduisait pas à de simples ajustements budgétaires d'ampleur modeste, comme on pouvait s'y attendre. Au contraire, il promeut en particulier l'une des nombreuses et foisonnantes mesures nouvelles que le Président de la République et son gouvernement égrènent au fil des semaines, à savoir l'indemnité inflation. J'y reviendrai. Certes, le Gouvernement bénéficie d'une très belle embellie économique, puisque les données de l'Insee publiées à la fin du mois d'octobre dernier montrent que l'activité s'est nettement redressée au troisième trimestre de cette année. notre économie a retrouvé son niveau d'avant-crise, mais cela n'est pas le cas pour toutes les branches ; il faudra y être attentif, notamment pour les secteurs du commerce, de l'hébergement-restauration ou encore du transport. Au regard des derniers développements conjoncturels, la prévision de croissance du Gouvernement, révisée à 6,25 % pour 2021, paraît particulièrement, voire excessivement prudente.

le Gouvernement n'a pas jugé bon de réviser sa prévision d'inflation, alors que celle-ci sera très vraisemblablement dépassée. Dans ce contexte de reprise économique et d'amélioration de la situation sanitaire, nos finances publiques restent marquées par les stigmates de la crise que notre pays vient de traverser.

Par exemple, les dépenses primaires, corrigées du coût de ces dispositifs, ont, à elles seules, augmenté de 41 milliards d'euros entre 2020 et 2021, soit le double par rapport aux mesures d'urgence et de relance.

Rendez-vous compte : à lui seul, le déficit budgétaire de l'État franchit le seuil des 200 milliards d'euros, pour atteindre 205 milliards d'euros en 2021, dont près de 24 milliards d'euros de crédits non consommés l'an dernier et reportés sur 2021.

rechercher l'explication du déficit. Cela est dû aux mesures nouvelles que le texte comporte, principalement l'indemnité inflation qui pèse à hauteur de 3,6 milliards d'euros sur le déficit de 2021, mais aussi la majoration du chèque énergie ou encore le plan de réduction des tensions de recrutement. Le niveau réel du déficit exécuté pourrait toutefois être significativement moins élevé, comme cela a été le cas l'an dernier, en raison des sous-consommations prévisibles, notamment sur les plans de relance et d'urgence. À ce titre, la commission des finances a adopté deux amendements tendant à supprimer respectivement un milliard d'euros sur la mission « Plan de relance » et 2 milliards d'euros sur la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », compte tenu des sous-consommations constatées, mais aussi des perspectives de consommation qui restent faibles sur les programmes visés d'ici à la fin de l'année. Même avec ces annulations, les crédits disponibles sur ces dispositifs permettront de couvrir les besoins au titre du chômage partiel ou du fonds de solidarité et ne remettront pas en cause le financement des investissements prévus par l'Agence des participations de l'État. Là encore, il s'agit de ne pas cautionner le matelas de crédits que conserve le Gouvernement, sans que cela soit véritablement justifié devant le Parlement. Parlement. Certaines autres mesures plus classiques de fin de gestion sont particulièrement coûteuses, à l'instar de l'enveloppe de 2 milliards d'euros alloués à France compétences pour assurer son financement, auquel

En revanche, nous constatons que, loin de limiter ses effets aux dernières semaines de l'année, ce collectif budgétaire engage les dépenses pour l'avenir. En effet, les ouvertures de crédits sont plus importantes en autorisations d'engagement, notamment pour le plan de relance, avec 2,3 milliards d'euros supplémentaires sans crédits de paiement, ou pour la mission « Travail et emploi ». Par ailleurs, loin des ambitions de réductions de 50 000 emplois de l'État durant le quinquennat,

ne profitent toujours pas au désendettement. C'est bien dommage et cela me paraît encore une occasion manquée ! Au-delà de ces considérations générales sur votre budget rectificatif, monsieur le ministre, c'est finalement votre proposition d'instaurer une indemnité inflation qui ne nous convainc pas. Cette mesure court-termiste est au mieux une réaction à la crainte d'un retour du mouvement des « gilets jaunes », au pire une mesure électoraliste de près de 4 milliards d'euros. Là encore, excusez du peu Cette aide forfaitaire de 100 euros, qui ne ressemble à aucune autre, serait attribuée à 38 millions de personnes, indépendamment de la composition de leur foyer ou de leur exposition réelle à la hausse actuelle des prix des carburants, qui est pourtant qui est pourtant à l'origine de cette mesure, de l'aveu même du Premier ministre. Telle qu'elle a été construite, cette disposition cumule les inconvénients : un ciblage insuffisant, des effets de seuil massifs des risques d'effets d'aubaine préjudiciables à son efficacité au regard du coût élevé qu'elle représente pour les finances publiques. Monsieur le ministre, comment justifier qu'un parent isolé ayant plusieurs enfants à charge et gagnant 2 100 euros net par mois

Enfin, cette disposition me semble créer un précédent dangereux pour la conduite de la politique budgétaire dans les mois et années à venir. À certains égards, ce que je qualifierai de « revenu universel d'un jour » témoigne d'une forme d'accoutumance à la dépense publique « quoi qu'il en coûte Pour toutes ces raisons, la commission des finances propose au Sénat de supprimer l'indemnité inflation. Pour autant, je vous rassure, nous sommes, tout comme vous, attachés à la préservation du pouvoir d'achat des ménages les plus exposés à une forte hausse des prix des carburants.

(FMI) ne préconise d'ailleurs pas autre chose dans son dernier rapport consacré à la France : « Face Il conviendrait de mieux cibler l'indemnité inflation. » C'est la raison pour laquelle, en lieu et place de cette indemnité, je propose de mettre en place, tout d'abord, une majoration exceptionnelle de 150 euros de la prime d'activité, qui bénéficierait à elle seule à 4,5 millions de foyers, couvrant près de 9 millions de personnes. Contrairement à l'indemnité inflation, ce dispositif ciblerait directement les travailleurs pauvres et modestes, qui sont les plus susceptibles d'être exposés à la hausse des prix des carburants, notamment ceux qui résident en zone rurale.

pour renforcer les aides financières, notamment les aides à la mobilité, qu'ils ont déjà la possibilité de verser aux chômeurs et aux jeunes en parcours d'insertion. En s'appuyant sur des dispositifs existants, notre proposition ne remet pas en cause l'objectif d'un soutien financier rapide

rectificative a été marqué par une très forte réévaluation du déficit attendu pour cette année, à hauteur de 9,4 % du PIB, principalement en raison de l'ampleur des crédits budgétaires reportés de 2020 sur 2021, dont la consommation était alors estimée à 28,8 milliards d'euros. Ces crédits devraient finalement être consommés à hauteur de 24 milliards d'euros, le déficit ayant été ramené à 8,4 % du PIB au mois de septembre dernier, chiffre désormais abaissé à 8,2 %. S'il est en amélioration, il reste cependant exceptionnellement élevé. Notre pays connaît pourtant un redémarrage de sa croissance, qui est désormais évaluée à 6,25 % du PIB. Le Gouvernement reconnaît lui-même que la croissance définitivement constatée

En tout état de cause, la prévision de recettes fiscales est en hausse de 18,6 milliards d'euros par rapport au niveau prévu au mois

Il nous est promis que les annulations font consensus et ne relèvent que de sous-consommations, de réserves de précaution ou de dispositifs non mobilisés, alors que les ouvertures de crédits couvrent un éventail de mesures nouvelles indispensables.

Au-delà de la pertinence de cet instrument pour répondre à la problématique du pouvoir d'achat des Français les plus modestes, sujet que M. le rapporteur général vient d'évoquer et dont

le mois de février 2022. ayant pour objet d'en modifier, plus ou moins discrètement et, pour tout dire, de moins en moins discrètement, les équilibres. La parole

rectificative prévoit d'annuler 135 millions d'euros en crédits de paiement, et les crédits non consommés sont d'environ 1 %, soit environ 100 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2021.

déficit public et de la dette publique » et que « le remboursement de la dette est une obligation impérative vis-à-vis des générations qui viennent, pour assurer la crédibilité française par rapport à ses partenaires européens et pour éviter d'avoir à dépenser de l'argent public afin de rembourser une charge d'intérêt

Pour autant, les dépenses nouvelles, qui, elles, sont certaines, sont compensées par des annulations de dépenses dont la réalisation était peu probable. Je pense ici aux crédits placés en réserve de précaution, à la réduction des appels en garantie ou encore aux dépenses accidentelles et imprévisibles, que le Gouvernement a provisionnées à hauteur de 1,5 milliard d'euros dans

Nous devons nous en féliciter, car ces formations participent à une meilleure employabilité des salariés. Cependant, France compétences est un organisme mal né.

Plus de 500 demandes restent à étudier, alors que la date butoir pour le renouvellement de l'enregistrement est fixée au 31 décembre 2021. Les professionnels du monde de la formation dénoncent une commission opaque dont les critères de décision sont complexes. en outre été surprise de constater, dans les décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux publiées le 10 novembre dernier, que des formations certifiantes en langue vivante comme le TOEIC,, sont accréditées pour un an seulement, quand des formations pour « réaliser des interventions sociales par le jeu de clown dans le secteur médico-social et dans l'événementiel » sont accréditées pour trois ans ou que des formations pour « préparer et animer une formation interne dans une entreprise de remontées mécaniques et domaines skiables » le sont pour deux ans.

À droite et au centre, nous nous interrogeons sur l'augmentation infinie de la dette de l'État, sur le poids qui pèsera sur les générations futures et sur le rôle de l'État, qui ne peut être un État nounou ou un État père Noël sortant son chéquier à chaque crise du pouvoir d'achat. un consensus se dessine : cette mesure, à quelques mois de l'élection présidentielle, est purement opportuniste. La politique du chèque n'a jamais permis de régler les problèmes de fond. Quel est le devenir de cette prime ponctuelle si, demain, les prix des carburants continuent d'augmenter ? 4 milliards d'euros pour la prime inflation, équivaut à quatre fois le montant consacré au nucléaire dans le plan France 2030 ! Avant d'entrer dans le détail de la mesure proposée, je tiens à faire un point sur le prix à la pompe. Le 15 octobre dernier, nous avons atteint un plus haut historique à 1,56 euro par litre en moyenne, soit 8 centimes d'euro de plus que le pic des mois de mars 2012 ou de novembre 2018. En d'autres termes, un plein coûte 4 euros de plus qu'il y a dix ans. Cette hausse n'est pas imputable au prix du baril.

payé par les consommateurs en 2008 et 2021 résulte pour partie de la hausse de la fiscalité verte, qui rapporte aujourd'hui plus de recettes à l'État que l'impôt sur le revenu. Les taxes sur le carburant ont augmenté de 16 centimes d'euro pour le gazole et de 4 centimes d'euro

La décision de verser cette indemnité est une nouvelle étape dans le dérèglement de notre politique économique. Cette disposition ouvre la voie à une société sous assistance permanente. Hier encore, je lisais un article sur la hausse du cours du blé. Demain, nous inventera-t-on un chèque baguette ?

En effet, au terme de cette année 2021, encore marquée par la crise, on constate que notre économie, et c'est tant mieux, a repris du poil de la bête.

Depuis, les lois de finances rectificatives se sont multipliées. Elles ont toutes été adoptées, même si elles comportent de nombreuses mesures fiscales et des mouvements de crédits qui ont considérablement affaibli nos travaux parlementaires.

Pour l'heure, il s'est cantonné à deux chèques symboliques de 100 euros ponctuels, qui s'apparentent déjà à des chèques préélectoraux. Rassurons-nous, l'indemnité inflation, remodelée par la majorité sénatoriale, et le chèque énergie n'aggraveront pas le déficit.

Pour le gaz, les distributeurs se rattraperont en maintenant leurs prix lors des futures baisses de cours- c'est le « lissage » des prix, version Jean Castex. Pour l'électricité, la baisse des taxes devrait être compensée par l'augmentation des dividendes versés par EDF à l'État. Le chèque énergie, lui, sera financé par les recettes de TVA supplémentaires liées à l'augmentation des prix avant le blocage. C'est donc un trompe-l'oeil, qui revient à faire payer le contribuable pour prétendument épargner le consommateur. Je vous rappelle, mes chers collègues, qu'une augmentation des prix, qu'elle figure sur une facture

Des choix politiques audacieux doivent répondre aux carences des dispositifs de court terme pris par le Gouvernement. Ce n'est pas aux Français de payer les dividendes des fournisseurs d'énergie

Nous proposons donc d'instaurer une contribution de 10 % sur les profits dégagés par ces fournisseurs sur l'année 2021. Quelle indignité de faire payer aux usagers des taxes sur les taxes de l'énergie La réponse à la précarité doit s'inscrire dans un programme structurel à long terme. Elle ne peut admettre comme seule réponse des distributions de chèques au gré des cours de marché. Vous le comprendrez, mes chers collègues : pour toutes ces raisons, et sans faillir à notre esprit de responsabilité, nous voterons contre ce projet de loi de finances rectificative.

d'un second projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours. Un tel schéma est habituel. À chaque fin d'exercice en effet, un budget rectificatif doit tirer les conséquences de l'année écoulée et proposer un schéma de fin de gestion.

Ces mesures peuvent se concevoir pour protéger les Français face à l'augmentation du coût de la vie, notamment du prix des carburants, de l'électricité et du gaz, qui accompagne la reprise économique observée en France et dans le monde. Elles n'en demeurent pas moins des réponses très ponctuelles, et très coûteuses, à un problème présenté, certes, comme temporaire, mais qui pourrait, hélas, durer encore de longs mois.

probablement pas continuer à sortir le chéquier bien longtemps ! Les membres du groupe Union Centriste, dans leur très grande majorité, ont pris leurs responsabilités. Nous avons salué et appuyé l'action du Gouvernement lorsqu'il s'est agi de soutenir les entreprises de notre pays, de sauvegarder l'emploi et à travers lui le tissu social, social, et lorsqu'il s'est agi, plus globalement, de maintenir à flot l'activité économique menacée d'effondrement devant la propagation du covid-19. Nous ne sommes pas naïfs pour autant. Si le déficit et la dette publics peuvent croître en période de récession, il est indispensable d'en reprendre aussitôt le contrôle, pour pouvoir garantir aux créanciers de l'État la signature de la France. Ce moment nous paraît venu.

nous vous proposerons deux amendements visant, respectivement, à orienter le surplus d'épargne « covid » vers les fonds propres des entreprises et à instaurer, en s'inspirant de l'exemple italien, une clause anti-abus

Aujourd'hui, malgré une hausse saisonnière des cas de covid-19, la nécessité d'inscrire des mesures d'aménagement face à la crise dans ce second projet de loi de finances rectificative pour 2021 ne relève pas de la même urgence, la vaccination à grande échelle ayant porté ses fruits.

Les principaux points à retenir sont les suivants. L'article liminaire tend à ramener le déficit budgétaire pour 2021 à 8,2 % du PIB, contre 8,4 % dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2022 ou encore 9,4 % dans la première loi de

L'article 1 majore la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour neutraliser certains mouvements financiers. Il s'agit de compenser le coût des dons de vaccins à des pays tiers et le transfert de ressources d'investissement du Ségur de la santé. plus de un milliard d'euros qui est transférée à l'assurance maladie. L'article 2 modifie les ressources du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » pour tenir compte d'une baisse de 160 millions d'euros liée à la chute du trafic routier.

Le déficit prévisionnel de l'État s'établirait donc en 2021 à 205 milliards d'euros, contre 220 milliards d'euros avec la première loi de finances rectificative pour 2021, soit une amélioration de près de 15 milliards

des agences régionales de santé ou encore de la Société de livraison des ouvrages olympiques. Quant à l'article 12, certainement le plus médiatique de ce projet de loi de finances rectificative, il instaure une indemnité inflation

Pourquoi ne pas aller plus loin en matière de redistribution ? Pourquoi ne pas faire davantage pour donner aux Français les plus modestes les moyens de vivre dignement dans un contexte encore très difficile ? Les leçons de la crise des « gilets jaunes » sont-elles déjà oubliées ? Avec le chèque énergie, l'indemnité inflation destinée à compenser la hausse des prix, notamment due à l'explosion des tarifs de l'énergie, est présentée par le Gouvernement comme le moyen de préserver le pouvoir d'achat de certains de nos concitoyens.

vaille, celui-ci continue de préserver d'abord les plus riches et avance une petite mesure pour tenter d'éteindre, à grand renfort de communication, la protestation sociale qui couve. D'ailleurs, on peut facilement comparer ce montant

qui cachent mal l'incapacité du Gouvernement à mesurer une réalité sociale et à mener une politique équilibrée. D'ailleurs, monsieur le ministre, vous aurez jusqu'au bout manqué l'occasion de créer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les hauts revenus ou sur les plus gros patrimoines. Même Nicolas Sarkozy

5,5 % pour agir vite et fort -, ainsi qu'un amendement tendant à accroître le montant du chèque énergie et à soutenir davantage les Français les plus modestes face à l'inflation.

Depuis deux ans, nous nous étions presque habitués à voter des budgets rectificatifs destinés à faire face à la dégradation des perspectives sanitaires et économiques. Aujourd'hui, la situation est différente l'amélioration des perspectives économiques et de nos finances publiques nous permet de retrouver un projet de loi de finances rectificative d'une autre nature, avec un déficit en net recul,

Il en découle des perspectives favorables pour nos finances publiques. Les recettes fiscales de l'État devraient être supérieures de 18,6 milliards d'euros au montant prévu lors de la précédente La situation de l'emploi est en nette amélioration, avec un taux de chômage désormais estimé à 7,6 %, soit le niveau le plus bas atteint depuis

La progression des indicateurs économiques pourrait encore améliorer ces chiffres d'ici à la fin de l'année. Ces bons résultats ne doivent rien au hasard ! L'État a été au rendez-vous durant toute la crise, comme nous l'avons tous constaté dans nos territoires. Le fonds de solidarité a bénéficié à plus de 2 millions d'entreprises et le chômage partiel à près de 9 millions de salariés. L'encours des prêts garantis par l'État a représenté un effort de 141 141 milliards d'euros au profit de près de 700 000 entreprises. Ces dernières ont également bénéficié de plus de 3,6 milliards d'euros de report de charges. La relance a permis une reprise rapide de notre économie au moment précis où les entreprises avaient besoin de remplir de nouveau leurs carnets de commandes. Ce sont ces choix forts qui nous permettent aujourd'hui d'annuler un certain nombre de dépenses d'urgence et d'améliorer d'autant l'équilibre de nos finances publiques. Je pense notamment à l'extinction du dispositif de prise en charge des coûts fixes. Au total, c'est une annulation de plus de 2 milliards d'euros sur la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », venant s'ajouter à la suppression de la dotation relative aux dépenses accidentelles et imprévisibles, qui a tant suscité d'émoi au printemps dernier et que le Gouvernement n'aura finalement pas eu besoin de mobiliser, faisant ainsi mentir ceux qui voulaient y voir un contournement de l'autorisation parlementaire. Cette autorisation sera amplement respectée, puisque l'exécution des dépenses ordinaires sera, en fin de compte, largement conforme aux prévisions de la loi de finances initiale. Nous pouvons d'ores et déjà dire que ce projet de loi de finances rectificative nous permet de respecter l'objectif de 5 % de déficit public en 2022.

Ce projet de loi de finances rectificative prévoit ainsi des ouvertures nettes de crédits de paiement pour un peu plus de 3 milliards d'euros au titre du relèvement exceptionnel de 100 euros du chèque énergie et de l'indemnité inflation. Ce sont au total 38 millions de Français, salariés, indépendants, retraités, chômeurs, allocataires des minima sociaux, étudiants boursiers, qui recevront 100 euros pour faire face à la flambée des prix, tant que leurs revenus ne dépassent pas le seuil de 2 000 euros.

le renforcement du fonds de stabilisation des départements, on peut dire que ce budget finance des priorités utiles à la relance et à la conduite de nos politiques publiques. Certains ont pu accuser le Gouvernement de « cramer la caisse Je m'étonne de ne pas les voir proposer la suppression de l'une ou l'autre de ces mesures. Peut-être en approuvent-ils, au fond, chacune des composantes ... Ces mêmes responsables politiques ne refuseront évidemment pas que l'État vole au secours d'Île-de-France Mobilités pour 800 millions d'euros cette année,

je l'ai indiqué en introduction, ce texte de fin de gestion recèle de nouvelles perspectives plus favorables qu'au printemps dernier. Cela permet de réduire largement le déficit, tout en apportant une réponse à la flambée des prix qui a touché tous nos concitoyens et que nous avons subie de façon particulièrement forte en outre-mer. sous-estime pour autant pas le chemin qu'il faudra parcourir pour redresser nos finances publiques. L'accord trouvé lundi soir sur la réforme du cadre organique des textes budgétaires nous invite à revoir les règles que nous nous sommes données voilà vingt ans. Il nous faudra pour les années à venir, quand la crise sera enfin derrière nous, réfléchir en profondeur à l'avenir que nous voudrons construire. La parole

dont l'article 6 crée une nouvelle catégorie de lois de finances : les lois de finances de fin de gestion. Cette nouvelle catégorie ne comporte aucune disposition fiscale. Elle se résume donc à de simples ajustements budgétaires de bonne gestion. Notre commission a salué cette initiative. C'était d'ailleurs la pratique du Gouvernement au cours des trois premières années du quinquennat. Sachant que cette mesure met pratiquement tout le monde d'accord, je souhaite partager avec vous deux interrogations. interrogation est la suivante : ce projet de loi de finances rectificative pour 2021 relève-t-il de cette nouvelle catégorie ? S'agit-il d'un texte technique, qui se résumerait à des opérations comptables de bonne gestion budgétaire ? La seconde interrogation découle de la première. Est-il souhaitable que ce texte relève de cette nouvelle catégorie ou faut-il encore voter des mesures d'urgence dans ce projet Pour tâcher de répondre à la première interrogation, je dirai que la plupart des mesures de ce texte n'appellent guère de commentaires. J'imagine, d'ailleurs, qu'elles ne feront pas vraiment débat.

Ils sont rendus possibles par l'embellie économique de cette fin d'année. Le rehaussement prudent de la croissance, à 6,25 % du PIB, et la baisse importante du chômage, désormais en deçà de son niveau d'avant-crise, ont conduit à une augmentation nette des recettes fiscales. Au global, le niveau du déficit s'établit à 5 %, bien plus près de la barre symbolique des 3 % de Maastricht que de celle des 10 % que nous avons franchie au plus fort de la crise. En clair, nous sommes sur la bonne voie pour sortir de cette crise. Bien sûr, je n'ignore pas l'avis du Haut Conseil des finances publiques, qui a recommandé de mettre à profit cette embellie pour désendetter le pays. Toutefois, cette recommandation va à l'encontre de toute la stratégie adoptée par la France pour lutter contre la crise sanitaire. loi de finances rectificative entre 2020 et 2021 pour mettre en oeuvre le « quoi qu'il en coûte ». Chacun peut bien penser, sous son masque, que la crise est terminée. Je crois pour ma part qu'il est sage de poursuivre cette année les mesures de soutien à l'économie, d'autant plus que l'épidémie semble réapparaître. Le Haut Conseil des finances publiques est certes d'excellent conseil, mais ce n'est pas à lui de prendre les décisions politiques. nous renvoie bien à des arbitrages d'ordre politique. Non seulement nous devrons décider si nous acceptons ces redéploiements de crédit, mais nous devrons aussi nous prononcer sur l'article 12, qui met en place l'indemnité inflation. Cet automne, alors que la hausse des prix de l'énergie faisait peser de lourdes incertitudes sur le pouvoir d'achat des ménages, les responsables politiques de tous les bords ont exhorté le Gouvernement à répondre à l'urgence. C'est chose C'est chose faite : désormais, la proposition est sur la table. Il ne nous reste plus qu'à en discuter les modalités. Faut-il cibler le dispositif sur les conducteurs de véhicules thermiques, plutôt que sur l'ensemble de la population ?

Il comporte de vraies mesures politiques, qui renvoient à une stratégie de sortie de crise sanitaire et à une volonté claire de soutenir les entreprises et les ménages. Pour le tout dernier projet de loi de finances rectificative du quinquennat, mon groupe aborde les débats avec sérénité.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

un projet de loi de finances rectificative de fin d'exercice est rarement l'occasion de discussions de fond très marquées. Ce texte traduit d'ailleurs, pour une grande partie, des ajustements classiques en la matière. Néanmoins, quelques remarques s'imposent. Si l'on peut se réjouir d'un niveau de croissance revu à la hausse, à 6,25 %, du fait d'une conjoncture économique très favorable, c'est avant tout la conséquence- certes, positive -de la sortie de crise, que nous espérons tous durable. cette croissance doit profiter à l'ensemble de la population. Or nous savons bien que, de ce point de vue, nous sommes loin du compte. Avec une inflation prévue à 1,5 %, principalement due au rebond des prix de l'énergie, le pouvoir d'achat de nos concitoyens déjà éprouvés par la crise va se trouver considérablement amoindri. Le Gouvernement nous assure que l'inflation sera compensée par la hausse des revenus. Cet argument est pour le moins trompeur, car il cache des écarts de revenus de plus en plus importants au sein de la population française, laquelle se répartit en trois catégories : les plus nantis, qui font l'objet de toutes les attentions, les classes moyennes, dont le pouvoir d'achat ne cesse de s'éroder, les plus précaires, qui sont les oubliés des politiques publiques de ce quinquennat. On m'objectera que tel n'est pas le cas, bien au contraire, en invoquant le chèque inflation. Qui peut, en cette fin d'année, s'opposer au versement de 100 euros aux Français gagnant moins de 2 000 euros par mois ? La réponse est évidente, mais le mécanisme n'en pose pas moins question.

Il faut dire que, pour l'État, les recettes supplémentaires de TVA sont considérables, avec la hausse des prix de l'énergie et du carburant. Actuellement, 25 centimes d'euros de TVA sont perçus par l'État sur chaque litre de carburant ; bien entendu, cette somme croît avec la flambée des prix à la pompe. J'avoue que, comme modèle d'économie circulaire, j'avais autre chose en tête qu'un recyclage de TVA ! De plus, cette aide fera l'objet d'un seul et unique versement. Elle ne traduit nullement la volonté du Gouvernement d'entreprendre une quelconque redistribution des richesses. loi de finances rectificative donne la priorité au désendettement au détriment de la cohésion sociale. Au-delà de la communication, le chèque inflation illustre la politique du Gouvernement : agir en faveur des plus aisés en maintenant l'illusion d'un accompagnement des plus fragiles. En effet, les fonds mobilisés sont relativement faibles en comparaison des cadeaux fiscaux faits aux très riches, Rémi Féraud en a parlé tout à l'heure. Parallèlement, rappelons que la baisse de l'aide personnalisée au logement (APL) n'a pas vraiment contribué à améliorer la situation financière des plus modestes

de retards, essentiellement liés à la crise sanitaire, concernant des projets immobiliers, soit d'un meilleur pilotage de certains postes- je pense notamment à l'aide juridictionnelle -, à la suite des travaux engagés par la Chancellerie.

je reviendrai également sur les plafonds d'emplois. Je précise d'ores et déjà que la prise en compte des mouvements opérés au cours de l'année 2021 ne remet pas en cause l'objectif, très actualisé- j'en conviens

Il n'est plus à prouver que le groupe communiste s'emploie à faire contribuer les personnes les plus aisées et les grands groupes afin de restaurer le consentement à l'impôt. Or, pour atteindre une réelle adhésion à l'impôt et aux taxes, il faut absolument en finir avec les taxes qui taxent des taxes.

200 millions d'euros sur le gaz et autant sur le fioul domestique. Sur une facture moyenne de chauffage, la « double peine fiscale » s'élève à 62 euros par an pour les ménages chauffés au fioul, à 56 euros pour les ménages chauffés

de l'électricité. Le Gouvernement a choisi de limiter cette hausse à 4 % : c'est un choix politique, d'autant que l'augmentation sera probablement lissée. Le phénomène d'augmentation des prix de l'énergie constitue une tendance de fond qui risque de s'accentuer à mesure que le mix énergétique inclura davantage de renouvelable. L'énergie nucléaire est moins chère, décarbonée et pilotable. Nous avons besoin de nucléaire et de renouvelable. Toutefois, des mesures pérennes doivent être prises pour limiter l'impact de cette transition progressive sur le montant des factures et,, sur le budget des ménages. Alors que le consentement à l'impôt a été gravement écorné par ce quinquennat,

Bref, supprimons les taxes sur les taxes pour ne pas ajouter de la précarité à la précarité !

supprimer la TVA sur les taxes, notamment la contribution au service public de l'électricité (CSPE), les taxes locales sur la consommation finale d'électricité (TLCFE) et la contribution tarifaire d'acheminement

de financer les aides exceptionnelles : à profits exceptionnels, taxes exceptionnelles ; à dépenses exceptionnelles pour les Français, aides exceptionnelles.

mettre à contribution les entreprises qui dégagent ces profits exceptionnels. Ainsi, nous répondrons à une inquiétude très souvent exprimée sur ces travées en luttant contre les déficits excessifs

pour la production nucléaire et hydraulique en France, qui bénéficie de prix de marché de l'électricité plus élevés ». En d'autres termes, les Français paieront non seulement l'envol des bénéfices des fournisseurs, mais aussi les mesures gouvernementales. a choisi, non seulement de ne pas toucher aux bénéfices des fournisseurs, mais aussi de rendre neutre en valeur le gel des tarifs du gaz en prévoyant des mesures de compensation. Selon nous, cette taxe interviendrait à un moment opportun. La Commission de régulation de l'énergie a mis en garde les fournisseurs alternatifs qui profitent de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh). On parle de rabais jusqu'à deux fois moins élevés que le prix de gros. Depuis l'ouverture du marché à la concurrence, en 2007, ces fournisseurs fixent leurs prix quasi librement. Les consommateurs qui ont fait appel à eux ne sont pas protégés contre une flambée des prix de l'énergie. Il était tentant, pour certains fournisseurs, de répercuter la hausse spectaculaire actuelle sur leurs clients.

? Ces amendements visent à créer une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé lors des six premiers mois de l'année 2021, par les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel et de carburant.

En 2020, ce groupe a versé 7,6 milliards d'euros de dividendes, malgré une perte nette consolidée de 7,3 milliards d'euros. Il perd de l'argent, mais verse des dividendes : allez comprendre ! Pis, cette entreprise a émis des obligations à hauteur de 15,8 milliards d'euros pour verser un dividende plus que généreux sur sa trésorerie.

le législateur s'est senti obligé de préciser : « Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. » Tel est le sens de cet amendement.

sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ? Les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions dont le régime et l'objet sont similaires à ceux des fonds de capital-investissement qui sont ouverts aux investisseurs non professionnels. Pour des raisons de structuration liées au fonctionnement des sociétés de capital-risque, les actions émises peuvent prendre la forme d'actions de préférence. Or ces actions sont exclues du champ des investissements éligibles aux PEA pour les particuliers, ainsi qu'aux PEA dédiés au financement des PME et des ETI. Introduire une exception de principe spécifique aux sociétés de capital-risque créerait un différentiel de traitement entre ces sociétés et les autres sociétés par actions, qui ne nous semble pas justifié. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'a pas changé d'avis depuis la loi de finances initiale : il reste défavorable

Ces bénéfices exceptionnels seraient calculés en comparaison de la moyenne des bénéfices réalisés dans les trois dernières années ou, à défaut, d'un taux de rendement de référence du capital.

les entreprises de la finance. BNP Paribas se félicite d'un bénéfice net « en forte hausse au troisième trimestre ». Le Crédit agricole annonce des résultats « à des plus hauts historiques ». Au troisième trimestre de 2021, la Société générale a même réalisé « le meilleur trimestre de son histoire

Il s'inscrit en cohérence avec les engagements du Gouvernement d'une compensation à l'euro près de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour les collectivités. En effet, la loi de finances pour 2020 a entériné et précisé les conditions et modalités d'application de la réforme de la taxe d'habitation, lancée en 2017, coopération intercommunale (EPCI) d'une compensation de leurs pertes de taxe d'habitation sur les résidences principales, sous la forme de l'attribution d'une fraction de TVA égale au produit résultant des bases de taxe d'habitation de 2020 et du taux de taxe Or le mode de calcul actuel de compensation de la suppression de la taxe d'habitation ne prend pas en compte, pour les EPCI créés en fusion à compter du 1 janvier 2018, la part de taxe d'habitation transférée des communes anciennement membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) vers le nouvel EPCI, issu de la fusion.

L'absence de prise en compte du mécanisme de « rebasage » de la fiscalité ménages dans les EPCI à fiscalité additionnelle conduit en effet à minorer artificiellement le taux 2017 de taxe d'habitation d'un EPCI issu d'une fusion

par des fusions d'EPCI à fiscalité professionnelle unique et d'EPCI à fiscalité additionnelle, occasionnant un rebasage entre les communes membres de l'ancien EPCI à fiscalité professionnelle et celles du nouvel EPCI à fiscalité professionnelle unique. Cela passe concrètement, vous l'avez indiqué, par une hausse de taxe d'habitation de l'EPCI, concomitante à une baisse de taxe d'habitation des communes concernées,

Monsieur le ministre,

DPEL est destinée à améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

critère d'éligibilité le potentiel financier par habitant, qui doit être inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permet une

ce qui ne me paraît pas pleinement justifié. Je relève d'ailleurs que des efforts importants ont été accomplis sur la DPEL, puisque, entre la loi de finances initiale de 2020 et celle de 2021,

la crise des scolytes, la baisse du nombre de locations de salles communales, et tout ce qu'elles ont dû vivre ... Certes, il s'agit de la dotation « élu local », je ne vais pas tout mélanger. Mais puisqu'on a permis la revalorisation des indemnités des élus locaux, il faut aussi accompagner les petites communes dans cette revalorisation.

masques, gel, gants, blouses -pour leurs employés, les bâtiments et les services sous leur responsabilité. Ainsi, certaines communes qui disposent de budgets modestes ont rencontré des difficultés financières. Plusieurs communes de mon département m'ont alerté sur la part importante de ces dépenses qui se sont ajoutées dans les budgets des années 2020 et 2021.

cofinancé par leur employeur pendant leur pause de travail contrainte par la journée continue. En 2021, plus de 4,5 millions de salariés bénéficient de ce droit social cofinancé par 140 000 employeurs privés comme publics et utilisé quotidiennement auprès de 220 000 restaurateurs ou commerces de proximité. Aujourd'hui, face à l'augmentation des prix des produits alimentaires de base et à sa répercussion sur les tarifs de la restauration, ce dispositif social nécessite quelques ajustements pour que les salariés accèdent à des repas de qualité. Ainsi le présent amendement vise vise à revaloriser le montant maximal de la participation patronale au titre-restaurant à 7,50 euros au lieu de 5,55 euros. Cela permettrait d'atteindre, avec la part de contribution du salarié, un plafond de 15 euros, qui correspond au prix moyen constaté d'un repas. Par ailleurs, afin de ne pas augmenter automatiquement le montant cofinancé par les salariés, il est proposé que la contribution ces derniers puissent être comprises entre 25 % et 50 % du prix du repas. Cette double mesure ne doit pas être assimilée à un coût pour l'État. En effet, le titre-restaurant n'est pas un salaire déguisé, qui échapperait à des cotisations sociales ou à l'impôt sur le revenu. Il est avant tout un droit social des salariés lié aux contraintes de travail, au même titre que les congés payés ou les remboursements de transport entre le domicile et le lieu de travail des salariés. Quel

Premièrement, il prévoit de déterminer dans la loi le montant des titres-restaurants cofinancés par les salariés, alors que cette disposition relève du domaine réglementaire. Deuxièmement, votre dispositif n'est pas borné dans le temps, contrairement à l'amendement que nous avions adopté lors de l'examen du premier projet de loi de finances rectificative

projet de loi de finances ou au début de l'année 2022, parce que la plupart des ceux qui regardent l'évolution des cours prévoient que les prix du pétrole vont continuer d'augmenter dans les prochains

je rappelle que, en application de l'article 42 de la loi organique du 1 août 2001 relative aux lois de finances et de l'article 47 , alinéa 2, du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances rectificative, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

résultat fortement déficitaire et un endettement qui devrait encore se dégrader pour atteindre, en 2021, plus de 508 millions d'euros.

Dans le contexte de crise énergétique que nous connaissons et qui se traduit durement sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, le chèque énergie exceptionnel mis en place par le Gouvernement n'est pas assez ambitieux ; il convient d'aller plus loin dans l'abondement du dispositif. C'est pour cela que cet amendement tend, en premier lieu, à ne pas annuler les crédits du programme 181, « Prévention des risques », et, en second lieu, à prélever ces crédits

Accompagnement transition énergétique, du programme 174, « Énergie, climat et après-mines ». Les auteurs du présent amendement précisent qu'ils ne souhaitent en aucun cas diminuer les crédits de l'Ademe,

le dispositif de prime à la conversion pour les transférer vers un programme qui « n'a rien à voir avec la choucroute », si vous me permettez cette expression, puisqu'il a vocation à financer le développement des infrastructures routières, principalement les

atteints par le covid-19 ... Prenant acte de ces difficultés supplémentaires occasionnées par la crise, l'éducation nationale a pris le parti de créer 1 500 ETP dès la rentrée 2021, pour renforcer l'accompagnement scolaire des élèves par la mise en place de plans d'accompagnement personnalisé. C'est une réponse indispensable au regard des enjeux.

la question spécifique du renforcement des moyens alloués à l'accompagnement scolaire n'a pas été prise en compte. Ainsi, une fois de plus, la logique de parité qui devrait prévaloir entre l'enseignement agricole et l'éducation nationale est « aux abonnés absents est d'autant plus regrettable que les conditions matérielles et humaines d'exercice, dans l'enseignement agricole, sont déjà extrêmement tendues, du fait des suppressions successives de postes depuis le début du quinquennat, dans un contexte général de réforme ne prenant pas réellement en compte les spécificités de cet enseignement.

pour un montant total de 2 853 900 euros. Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il a été nécessaire de le gager, mais nous demandons au Gouvernement de lever le gage. Quel est l'avis de la commission loi de finances rectificative prévoit déjà l'ouverture d'un peu plus de 8 millions d'euros pour les établissements de l'enseignement technique agricole en difficulté, afin notamment de recruter des assistants d'éducation supplémentaires.

disponibles. Les crédits ouverts pour 2021 et non encore consommés à ce jour sur le programme 364 permettent de faire face à nos engagements et ne remettent pas en cause l'équilibre budgétaire.

monsieur le ministre,

jusqu'à la fin de l'été dernier, nous avons maintenu un régime de financement de l'activité partielle à un niveau extrêmement élevé, ce que tout le monde a salué, parce que cela préservait les emplois et la majeure partie des revenus.

Voilà pour les nouvelles peu réjouissantes concernant ce dispositif innovant, adopté, je le répète, à l'unanimité de la Haute Assemblée. Revenons-en au présent texte. Durant la crise, ces associations, comme des milliers d'autres associations de solidarité, se sont révélées être d'indispensables amortisseurs sociaux : fabrique de masques, distribution d'objets et de nourriture aux plus vulnérables, continuité du travail social.